d’observation ?… Le procès verbal est adopté sous les réserves d’usage. Madame la Première ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l’ordre du jour appelle les questions d’actualité au Gouvernement.

jours de violation du droit international. Trente jours où, sous couvert de combattre le terrorisme, on le nourrit et le renforce ; Dominique de Villepin le rappelait hier encore, ni la force ni la vengeance n’assurent la paix et la sécurité : seule la justice peut le faire. jours que nous attendons une parole forte et claire de la France, pour un cessez le feu, le retour de l’aide humanitaire et la libération des otages ! Le soutien inconditionnel de la France aux opérations militaires d’Israël et à l’occupation est une erreur tragique, qui marquera l’histoire de façon dramatique. Cela ne sert ni les Israéliens ni les Palestiniens. Depuis dix ans, la France a vendu pour 209 millions d’euros d’armes à Israël – des bombes, des roquettes et des missiles utilisés contre la population de Gaza. La France a pourtant ratifié le traité sur le commerce des armes de l’ONU, dont l’article 6 impose l’arrêt des transferts d’armes si celles ci sont employées pour commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des attaques dirigées contre des civils ou des crimes de guerre.

Comptez vous adopter un embargo sur les ventes d’armes, comme l’avait fait le général de Gaulle lors de la guerre des Six Jours ? Comptez vous reconnaître l’État palestinien, comme le Parlement l’avait voté en 2014 ? Comptez vous appeler à l’arrêt et au retrait des colons pour préserver la solution à deux États ? Madame la Première ministre, face à cette folie meurtrière, nous avons besoin de réponses précises. de réponses précises. La parole est à Mme la Première ministre. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Guillaume Gontard, depuis les terribles attaques terroristes perpétrées par le Hamas contre Israël, la situation dans la région est extrêmement préoccupante. Israël a le droit d’assurer la sécurité de son territoire, mais cela doit se faire dans le respect du droit international, et nous devons impérativement éviter l’escalade et l’embrasement dans la région. Je le dis sans ambiguïté, la situation humanitaire dans la bande de Gaza est dramatique. Le bilan humain est extrêmement lourd, avec de nombreuses victimes civiles, notamment des femmes et des enfants. Les populations palestiniennes ne doivent pas payer pour les crimes du Hamas. Elles doivent être protégées de toute urgence. Cette urgence, la France n’a cessé de la réaffirmer, et nous avons condamné très clairement les frappes contre les personnels humanitaires et les sites de l’ONU. Comme nous l’avons dit, le droit international humanitaire impose des principes clairs de distinction, de nécessité, de proportionnalité et de précaution. La protection des civils est à la fois un impératif moral et une obligation internationale. Une trêve humanitaire immédiate et durable est absolument nécessaire. Elle doit pouvoir mener à un cessez le feu. Monsieur le président Gontard, la France est mobilisée pour la paix. Sur l’initiative du Président de la République, une conférence humanitaire internationale pour la population civile de Gaza se tiendra demain à Paris. J’ajoute que nous suivons de très près la situation de nos ressortissants dans la bande de Gaza. Nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de revenir en France ; plus de cent d’entre eux ont pu quitter Gaza depuis vendredi dernier. De plus, nous restons mobilisés pour obtenir une libération immédiate et sans condition des otages. Monsieur le président Gontard, face à ce conflit, la seule issue possible est une solution politique avec deux États. C’est la position invariable de la France. C’est le sens de l’initiative pour la paix et la sécurité pour tous que porte le Président de la République. Cette initiative la sécurité, avec une lutte implacable contre le terrorisme ; le soutien humanitaire, avec une réponse internationale rapide et forte face à l’urgence à Gaza la détermination à relancer un processus politique permettant de garantir à la fois la sécurité d’Israël et la création d’un État pour les populations palestiniennes.

il est tout à fait vrai qu’il y a en France une explosion du nombre des actes antisémites. Ces faits étaient déjà nombreux avant l’attaque terroriste du Hamas contre la population israélienne.

effet, à la demande du Président de la République et de la Première ministre, dès le premier jour, dans les 950 lieux où les Français de confession juive ont l’habitude de mener leurs enfants à l’école, vivre leur culte, ou simplement de vivre, nous avons mobilisé quasiment 11 000 policiers, gendarmes et militaires de l’opération Sentinelle, qui ont pu protéger ces Français contre de très nombreux actes antisémites et interpeller des personnes qui voulaient passer à l’acte.

une quarantaine d’entre eux sont en centre de rétention administratif. Nous avons déjà commencé les éloignements, comme vous avez pu le voir, parce qu’on ne peut pas toucher un Français de confession juive, un juif en France, sans toucher toute la République.

Merci

il faut accepter d’identifier sans tabou ses origines et ses ressorts. L’antisémitisme déguisé en compassion pour les Palestiniens se nourrit du wokisme et de sa haine de la culture occidentale. Dans ce domaine comme dans tant d’autres, Dans ce domaine comme dans tant d’autres, il n’y a pas de place pour le « en même temps ». Oui, il y a une culture française, qui puise ses valeurs dans notre histoire judéo chrétienne.

La vérité est que nous avons, sous couvert de tolérance ou d’accommodements dits « raisonnables », renoncé à notre identité et à notre culture pour épouser un relativisme culturel qui montre aujourd’hui ses limites et ses effets délétères.

L’antisémitisme, c’est la mort, entendez vous, de la civilisation européenne. » Des propos qui sont bien d’actualité… La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

Trois personnes ont perdu la vie – dans l’Aisne, au Havre et à Pont Aven, dans le Finistère, où Frédéric Despaux, employé d’Enedis, est décédé en intervention. Je souhaite également souligner le remarquable travail du préfet du Finistère et, à travers lui, saluer l’ensemble de la chaîne de secours et les services de l’État. Grâce au déclenchement du dispositif FR Alert et à la sensibilisation des populations en amont, des vies ont probablement été sauvées. Je n’oublie pas la formidable implication de nos élus et de nos agents territoriaux. Qu’ils en soient, dans cet hémicycle, remerciés vivement

particulièrement dans le secteur agricole, où des serres ont été écrasées, des bâtiments, parfois anciens, dégradés, et des éleveurs privés d’eau et d’électricité. La profession évalue le préjudice pour la ferme finistérienne à près de 200 millions d’euros.

L’afflux massif de mineurs isolés étrangers sur le territoire français constitue un véritable casse tête pour les départements, qui assurent la protection de l’enfance, même si ceux ci ont conscience que cet exode reste dramatique pour la plupart de ces

Les structures d’accueil sont saturées, malgré les efforts des départements pour dégager de nouvelles solutions d’hébergement spécialisé. De plus, la loi relative à la protection des enfants, dite loi Taquet, interdit à partir de 2024 l’hébergement dans des hôtels de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance

Madame la ministre, les départements demandent la mise en œuvre de deux mesures : d’une part, le transfert à l’État de la compétence de mise à l’abri des personnes se présentant comme mineurs non accompagnés, le temps de l’évaluation de leur minorité par le département ; d’autre part, la compensation à l’euro près des dépenses engagées pour la prise en charge des mineurs non

est pris en charge dans les mêmes conditions que les enfants de nationalité française. Depuis 2016, l’État soutient les départements, par un dispositif de répartition équilibrée des mineurs non accompagnés sur le territoire, mais aussi par une aide financière visant à compenser une partie des coûts qu’entraîne leur prise en charge.

le Gouvernement a lancé une enquête flash pour faire un état des lieux des difficultés de prise en charge rencontrées par les départements et en tirer les leçons. Sur cette base, avec Charlotte Caubel, Gérald Darmanin et Éric Dupond Moretti, autour de Mme la Première ministre, nous travaillons à des solutions de moyen et de long terme. Nous ferons tout pour trouver un consensus avec les départements. C’est sur la base de cette mission et dans la concertation avec l’ensemble des acteurs que nous pourrons prendre des mesures pertinentes. Il s’agit d’enfants ; notre mobilisation est totale et entière.

Déjà, le secteur du bâtiment, qui représente 6 % du PIB, 1 273 000 salariés et 403 400 entreprises artisanales, en ressent les répercussions. Les chiffres sont alarmants

Monsieur le ministre, il faut agir rapidement, car le secteur du bâtiment est un paquebot : beaucoup de temps s’écoule entre le moment où l’on remet les moteurs en route et celui où le navire retrouve sa vitesse de croisière. dans cette situation, vous supprimez le dispositif Pinel et vous écartez nombre de communes du nouveau prêt à taux zéro (PTZ). Une fois de plus, ce sont les territoires ruraux, supposés hors tension, qui sont oubliés. Pourtant, les besoins en logement y sont énormes et l’accès à la propriété y est un fort facteur d’attractivité.

C’est pourquoi je vous demande que les zones rurales soient éligibles aux nouvelles conditions du PTZ. Ainsi, vous assurerez l’attractivité du monde rural, qui, sans cette décision, continuera, encore et toujours, à se désertifier.

En zone tendue, là où il faut absolument construire de nouveaux logements, nous avons souhaité le concentrer sur le neuf, avec davantage de publics éligibles et une aide renforcée. En zone

Dans le Cantal, il y a 43 % de passoires thermiques et un taux de vacance de 12 %. Vous comprenez évidemment que, dans ces territoires, il nous faut privilégier l’aide publique destinée à l’acquisition rénovation.

Madame la Première ministre, cela fait cinq semaines que les Françaises et les Français dressent l’oreille. Ils sont inquiets, horrifiés, scandalisés par la résurgence de l’antisémitisme en France. Pas un jour ne passe sans que notre pays connaisse une nouvelle agression, une nouvelle menace, une nouvelle dégradation, une nouvelle mise en cause contre nos compatriotes de confession juive. Cette réalité là nous scandalise. L’antisémitisme, qui n’a jamais disparu de la société française, redouble d’acuité. Il s’étale sans complexe. Il menace, il sévit, il empoisonne la vie de nos concitoyens, de nos compatriotes. Madame la Première ministre, toutes les forces politiques républicaines et démocratiques se mobilisent, se dressent – votre gouvernement aussi. Le Président du Sénat et la Présidente de l’Assemblée nationale ont appelé à une manifestation dimanche prochain. C’est une heureuse initiative. Merci, monsieur le président Madame la Première ministre, nous avons besoin de savoir quelle est la genèse de ces faits, quels moyens sont mobilisés pour les empêcher et quelle est la volonté du Gouvernement de lutter contre la résurgence de l’antisémitisme, afin que chacune et chacun d’entre nous prenne sa part, toute sa part, sa juste part, dans la

collectivement, réfléchir à notre accès à ces plateformes. Quand 75 % des contenus antisémites signalés à la police viennent de Twitter, le ministre de l’intérieur se dit que les policiers ne peuvent pas tout faire : tout le monde doit prendre sa part.

Quatre mois après ces tragiques événements, la présentation du plan du Gouvernement était très attendue. Madame la Première ministre, vous avez dévoilé vos propositions il y a bientôt deux semaines, dans l’amphithéâtre de la Sorbonne. J’y étais, et je peux vous assurer que de nombreux élus en sont ressortis déçus. Vos propositions restent largement insuffisantes pour répondre aux enjeux de nos territoires. Votre plan mêle le tout répressif et le contrôle social ; il s’impose, telle une double peine, notamment aux familles monoparentales. Madame la Première ministre, avez vous bien entendu ce que demandent les élus locaux ? Ne pensez vous pas que, si des communes ont développé des polices municipales et demandent aujourd’hui leur armement, c’est tout simplement parce que les forces de l’ordre ont purement et simplement disparu de leur territoire ? Ne pensez vous pas que le triptyque prévention répression insertion gagnerait à ce que l’État assume clairement ses compétences régaliennes liées au maintien de l’ordre public ? À ce sujet, que proposez vous pour la prévention spécialisée, si utile pour nos quartiers ? Enfin, madame la Première ministre, parler de police de proximité, c’est parler de complémentarité.

nous développerons également des dispositifs visant leur insertion dans une vie citoyenne et active, comme les classes de défense ou le service militaire volontaire. qui concerne l’usage des réseaux sociaux – vous n’ignorez pas qu’ils ont joué un rôle de catalyseur dans ces émeutes –, nous créerons une peine complémentaire de suspension de compte utilisateur en cas d’infraction commise sur une plateforme en ligne.

pour le groupe Les Républicains. Ma question s’adresse à Mme la Première ministre. Nous sommes entrés dans une ère où la compétition stratégique entre les puissances est désormais la norme, et où la lutte contre les ingérences étrangères est devenue une préoccupation de chaque instant. La délégation parlementaire au renseignement en a d’ailleurs fait le thème central de son dernier rapport. Son président, Sacha Houlié, membre de votre majorité, madame la Première ministre, y propose un plan d’action pour protéger les intérêts économiques et scientifiques de notre pays. En résumé, il vous invite à sortir du déni. C’est un vœu similaire que nous formulions le 2 août dernier, avec mes collègues du groupe Les Républicains, dans une tribune intitulée : « Cessons de vendre nos fleurons les plus stratégiques à des puissances étrangères. Nous alertions sur la décision du groupe Atos de céder une partie de ses activités à la société EP Equity Investment, propriété du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Depuis cette publication dans les colonnes du, pas une semaine ne se passe sans un nouveau rebondissement chute vertigineuse du cours d’Atos, fronde des actionnaires, plaintes déposées auprès du parquet national financier (PNF), départ forcé du président d’Atos, ou encore, cette semaine, arrivée très opportune d’un nouvel investisseur. Bien sûr, Atos est une entreprise privée, mais elle n’est pas une entreprise comme les autres. C’est sur elle, sur ses supercalculateurs, que repose une partie de notre souveraineté nucléaire. Son démantèlement et, surtout, l’immixtion d’acteurs étrangers, fussent ils européens, dans son activité font peser un risque inacceptable. Alors que l’enjeu est crucial, comment comprendre le silence assourdissant de votre gouvernement sur cette question ? Madame la première ministre, reprenez les choses en main ! Le projet de M. Kretinsky fera t il, oui ou non, l’objet d’un contrôle au titre des investissements étrangers en France ? Nous attendons une réponse claire.

qu’une influence très marginale sur la vie de l’entreprise. Par ailleurs, nous n’hésiterons pas à activer le contrôle des investissements étrangers en France. Comme vous le savez, monsieur le sénateur, le code monétaire et financier soumet toute prise de participation par un acteur étranger dans une entreprise d’importance stratégique en France à une autorisation du ministre de l’économie et des finances. Et que fera t il ? Où est il ? Soyez assuré que, sous l’autorité de la Première ministre, le Gouvernement est attentif à l’avenir d’Atos comme à la garantie de la souveraineté numérique de la France. Monsieur le ministre, ceux qui, comme moi, attendaient une réponse claire en sont pour leurs frais ! De fait, l’absence de réponse à ma question obligera le Sénat à exercer son devoir constitutionnel de contrôle.

Hier soir, le Sénat a voté sa suppression, sans opposition de votre Gouvernement. C’est une digue de plus qui vient de sauter. Cette suppression s’est faite sur fond de cacophonie gouvernementale. Le 7 octobre dernier, M. le ministre Darmanin se déclarait favorable à la suppression de l’AME.

Ce mardi, ici même, après avoir prononcé un plaidoyer émouvant, ou presque, pour l’AME, après avoir indiqué l’attachement du Gouvernement à ce dispositif, après avoir marqué son opposition à la droite sénatoriale, Mme la ministre Firmin Le Bodo s’est totalement dédite en émettant un avis de sagesse, synonyme de blanc seing pour cette même droite sénatoriale. Le soir même, son ministre de tutelle, M. Aurélien Rousseau la désavouait, en regrettant cette suppression, qu’il qualifiait de « grave erreur ». Nous partageons l’avis de votre ministre – je Nous nous élevons contre cette posture politicienne de la droite sénatoriale, prête à sacrifier la santé des étrangers et les enjeux de santé publique dans un calcul électoral cynique. L’ensemble du corps médical est révolté. Nos hôpitaux s’en trouvent fragilisés. Une certaine idée de la République sociale est bafouée.

loi vise à atteindre un double objectif : d’une part, éloigner plus rapidement ceux qui n’ont pas vocation à rester sur notre sol ; d’autre part, mieux intégrer ceux que nous choisissons d’accueillir. ! Vous m’interrogez spécifiquement sur l’AME. Ma position est sans ambiguïté. C’est celle de mon gouvernement et elle a été exprimée très clairement hier. L’AME est un dispositif nécessaire, qui répond à un impératif de santé publique. Elle doit permettre de soigner les personnes malades qui sont sur notre sol. Elle constitue aussi une protection pour l’ensemble de nos concitoyens, car elle permet de prévenir la propagation de certaines maladies. Et contre la peste La prise en charge, au plus tôt, des infections respiratoires, des hépatites ou encore du VIH est une nécessité. Je veux ensuite souligner que l’AME est un dispositif très encadré et surveillé. C’est même le dispositif le plus contrôlé de l’assurance maladie. Pour débattre de ce sujet, nous avons besoin d’un diagnostic précis, objectif et actualisé.

est à Mme Françoise Dumont, pour le groupe Les Républicains.

n’a pas été rendu public. Pourtant, des journalistes ont pu s’en procurer un exemplaire… Dans ce document, il serait indiqué que, l’année dernière, les commissariats avaient à leur charge un stock ancien de 2,7 2,7 millions de plaintes ; un tiers d’entre elles seraient en stock depuis plus de deux ans. Il faudrait y ajouter 3,5 millions de nouvelles plaintes enregistrées dans le courant de l’année. Il y serait aussi indiqué que, en moyenne, un policier doit traiter 180 dossiers par an. Pour les enquêteurs les plus spécialisés, on parle de 800 dossiers Le rapport préciserait que « des dossiers portant sur des faits graves dorment dans certains services sans avoir fait l’objet d’investigations alors même que les auteurs présumés ont été identifiés ». continuer à augmenter d’ici à 2030 et passer à 3,5 millions de plaintes en attente. Dans un État de droit, il n’est pas possible de laisser des coupables dehors, en toute impunité. Dans un État de droit, il n’est pas possible de ne pas répondre au devoir de justice vis à vis des victimes.

avant la fin des délais de prescription des éventuels actes, passibles de sanctions pénales, visés par les quelque 2,7 millions de dossiers en souffrance ? La parole

le 22 mars dernier, le ministre de l’économie et des finances annonçait publiquement son intention d’interroger le Conseil d’État sur un possible raccourcissement de la durée des contrats de concession d’autoroutes.

ou une taxation – des sociétés autoroutières à notre stratégie de décarbonation et à notre plan d’investissement pour les transports. Sur le premier point, comme sur l’ensemble de ces questions, je suppose, les sociétés d’autoroutes ont déposé un contentieux.

Cela n’a pas été le cas : le Conseil d’État n’a pas décidé de suspendre ses travaux consultatifs. Il a rendu un avis que nous avons décidé, avec la Première ministre, de rendre public rapidement, dès la fin de

aucune autre suite judiciaire à ces événements, pas même pour ceux de L’Haÿ les Roses. Les émeutes qui se sont déroulées dans notre pays ont occasionné, d’après les assureurs, 650 millions d’euros de dégâts. Un millier de bâtiments publics ont été touchés. Ce sont les symboles de notre République qui ont été visés

objectifs auxquels je ne peux que souscrire. Selon les chiffres communiqués par le Gouvernement au cours de l’été, 1 000 condamnations ont été prononcées, principalement à de courtes peines, pour 10 000 émeutiers. Mais où en est on aujourd’hui ? La représentation nationale est en droit de disposer d’un bilan, département par département, du nombre de personnes interpellées et de personnes condamnées, avec le détail des peines et de leur exécution. Le garde des sceaux peut il nous confirmer que tous les moyens de l’État sont encore mobilisés pour mener les enquêtes, sanctionner les vrais coupables, les donneurs d’ordre, responsables de toutes les atteintes graves aux personnes et aux biens perpétrées durant ces quelques jours ? Il y va de la crédibilité de l’État et de celle des élus.

Le 30 juin 2023, le garde des sceaux a adressé une circulaire aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, afin qu’une réponse pénale rapide, ferme et systématique soit apportée à l’encontre des auteurs de ces exactions. Le traitement judiciaire de ces affaires a été effectif et empreint de célérité : un taux de réponse pénale de 92 %, un taux de poursuite par défèrement de 90 %. Le recours à la comparution immédiate a été massif, représentant 60 % des poursuites devant les tribunaux correctionnels. Près de 1 800 personnes ont été condamnées à une peine d’emprisonnement ; le quantum de peine moyen avoisine les neuf mois de prison ferme. Le ministre de la justice défend douze mesures concrètes visant à renforcer la répression envers les plus jeunes et à responsabiliser leurs parents.

un partenariat renforcé avec l’armée pour suivre certains mineurs délinquants, la création d’une responsabilité civile de plein droit pour les deux parents d’un mineur, même s’ils sont séparés,

Madame la Première ministre, la tempête Ciaran a très durement éprouvé la Bretagne. Il faut tout d’abord saluer l’engagement exceptionnel des pompiers, des agents des forces de l’ordre et de la sécurité civile, de ceux des collectivités territoriales, mais aussi de ceux des opérateurs, en particulier d’Enedis. Honorons la mémoire des victimes et rendons hommage à Frédéric Despaux, agent d’Enedis décédé dans l’exercice de ses fonctions. Nos pensées vont à sa famille et à ses collègues éplorés. Le monde agricole est très lourdement touché. Une réunion du comité catastrophe naturelle a été annoncée pour le 14 novembre, soit deux semaines après le début de la tempête : c’est bien tard

des élus ont dû utiliser leur propre véhicule pour aller chercher des groupes électrogènes, envoyés en Bretagne trois jours après le début de la tempête ; enfin, un maire a été obligé de faire six relances différentes en six jours pour mettre en sécurité deux points critiques. « Perdus au milieu de nulle part », pour reprendre leurs termes, obligés d’endosser des responsabilités majeures sans disposer des bonnes informations et des moyens appropriés, les maires et les élus sont à bout. La sous traitance de l’État confine désormais à la maltraitance. Nous voyons là les effets directs du désarmement de nos services publics, du sous investissement chronique et de la logique du flux tendu, qui ne nous permettent pas de faire face aux épreuves d’un monde qui se dérègle. Face à la multiplication prévisible des catastrophes climatiques, il est urgent d’agir. Quelles actions concrètes allez vous mettre en œuvre pour que cette situation ne se reproduise plus ?

rappeler que les dommages causés par les vents violents sont couverts par la garantie tempête des polices d’assurance souscrites par les collectivités, en vertu de l’article L. 122 7 du code des assurances.

est quand même très court, monsieur le sénateur ! Le décret paraîtra dans les jours qui suivront. Ce mécanisme bénéficiera évidemment aux collectivités territoriales et permettra, notamment, de couvrir les dommages liés aux phénomènes de submersion ou de de débordement des cours d’eau. Si des difficultés survenaient avec les assureurs quant au remboursement des dommages, nous ferions le nécessaire avec le médiateur des assurances, dont vous savez qu’il peut, depuis le mois de septembre, être saisi par les collectivités elles mêmes. Nous disposons enfin de la dotation de solidarité en faveur de

puissent être rapides et significatives. J’y veillerai personnellement. Par ailleurs, le ministre de l’agriculture poursuit les travaux d’évaluation des dégâts, afin d’enclencher toutes les procédures de reconnaissance de calamité agricole dans les délais les plus courts. Les pertes de récoltes seront prises en charge dans le cadre du nouveau système assurantiel, y compris pour les agriculteurs non assurés, par le biais de l’indemnité de solidarité nationale. Comme chaque fois, nous serons, bien entendu, aux côtés des collectivités, des agriculteurs et de tous nos concitoyens. La parole est à Mme Agnès Evren, pour le groupe Les Républicains.

Votre position a été courageuse : parents, enseignants, victimes, tous avaient besoin d’entendre ce message clair. L’omerta était devenue insupportable.

près de 80 % des parents se disent inquiets. Il y a donc urgence. Les faits, je le rappelle, sont sans précédent. Auparavant, le harcèlement scolaire s’arrêtait aux grilles de l’école, à seize

Ces moyens seront ils suffisants ? En effet, trop d’établissements gèrent la pénurie : celle des médecins, des psychologues, des infirmières scolaires. Pouvez vous nous confirmer que tous les personnels scolaires seront désormais systématiquement formés pour prévenir et détecter Allez vous rendre obligatoires les questionnaires d’autoévaluation, alors que les deux heures de temps scolaire banalisées sont facultatives ? Enfin, en matière de sanctions, pouvez vous nous donner des précisions sur la mise en place des mesures d’éloignement du harceleur

Ce fléau est absolument insupportable : des élèves vont à l’école la boule au ventre, parfois ils se donnent la mort, parce qu’ils subissent des brimades, des insultes, des coups.

les trois élèves harceleurs, âgés de 15 et 16 ans, ont été interpellés par les forces de police et placés en garde à vue. Ils passeront devant le juge des enfants le 15 novembre et ont d’ores et déjà été exclus de l’établissement. Comme eux, plusieurs dizaines de jeunes harceleurs ont déjà été exclus de leur établissement depuis que j’ai pris cette décision.

la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a estimé que la France ne peut pas procéder au refoulement vers un pays voisin d’une personne migrante entrée illégalement sur le territoire sans que celle ci puisse bénéficier d’un certain délai pour le quitter volontairement. Cet arrêt se

court circuite le droit national et nos procédures administratives, dans un contexte où la gestion des flux migratoires est très problématique. Je le constate dans mon département, les Hautes Alpes, où les migrants passent régulièrement entre l’Italie et la France, notamment les cols de l’Échelle ou de Montgenèvre.

monsieur le ministre. Nous attendons donc la décision du Conseil d’État. Je me permets d’appeler votre attention sur deux points relatifs à la frontière avec l’Italie dans mon département.

et à la décentralisation a été publiée. Cette candidature sera ratifiée si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. L’ordre du jour appelle la désignation des vingt trois membres de la commission d’enquête sur l’impact du narcotrafic en France et les mesures à prendre pour y remédier. En application de l’article 8 , alinéa 5, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 58 1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et du chapitre XVII de l’instruction générale du bureau, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration

renvoyés à leurs origines et à la nationalité de leurs parents, bien que la France soit le seul pays qu’ils aient connu de toute leur vie. On leur dit qu’ils devront toujours prouver qu’ils méritent d’être Français.

ajouter à ce que vient de dire Corinne Narassiguin, dont je partage pleinement les propos, que derrière cette « manifestation de volonté » que cherche à imposer la droite sénatoriale pour les jeunes arrivant à l’âge de 18 ans se cachent

cette disposition, adoptée par le Sénat en commission, devait subsister, on ajouterait une condition pour l’accès à la nationalité française d’un enfant né en France de parents étrangers. Celui ci devrait « manifester la volonté » d’acquérir la nationalité française. En d’autres termes, l’accès à la nationalité française pour ces enfants et adolescents qui n’ont, le plus souvent, pas connu autre chose que la France cesserait d’être automatique. Notre commission a donc décidé de faire renaître les lois Pasqua.

Je ne pense pas qu’une formalité administrative dise véritablement quelque chose de l’attachement à la France d’une personne. C’est également une question de principe : nous sommes attachés à la reconnaissance du droit du sol par notre nation.

du sol. Le code civil dispose aujourd’hui que tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle

De plus, nous craignons que des personnes n’ayant pas eu accès à cette information avant leur majorité, ou n’ayant pas réalisé l’importance de cette démarche pour leur avenir, se voient privées de leur nationalité – je rappelle que cette démarche devrait être faite entre l’âge de 16 et de 18 ans.

Il faut bien le dire, le combat de la droite française pour restreindre le principe du droit du sol n’est pas nouveau. On peut même parler d’une idée fixe. C’est reconnu ! Après la mise en place de la commission Marceau Long par le Premier ministre Jacques Chirac, c’est le gouvernement d’Édouard Balladur qui supprima l’automaticité du droit du sol pour les jeunes de 18 ans nés en France et y résidant depuis une certaine période. Le droit du sol, manifesté par la naturalisation de ces jeunes qui ont vocation, par leur lieu de naissance et leur résidence, à devenir Français, accompagne toute l’histoire de la République de 1851 à 1927, en passant par la loi de 1889, le droit du sol s’est ancré dans l’histoire de la République. Ce n’est pas vrai ! Faut il rappeler – nous le verrons avec les amendements de Mme Boyer,

! Comment ne pas se rappeler que c’est le gouvernement de Vichy qui inaugura l’idée de la remise en cause du droit du sol, avec la mise en place d’une commission de révision de naturalisation, triste instance qui doit encore faire rêver certains partisans de Mme Le Pen ou de M. Zemmour ! C’est l’ordonnance du 19 octobre 1945, issue du combat, main dans la main, des Français et des immigrés contre l’occupant nazi, qui instaura le droit du sol qui s’applique aujourd’hui dans notre pays. Nous n’acceptons pas la demande dangereuse de la droite sénatoriale, qui, au moment où la cohésion sociale de notre pays est menacée, décide de faire planer le doute sur l’avenir de toute une jeunesse. Le droit du sol a une origine, une histoire. Il a supplanté le droit du sang. Et rappelez vous qu’il fut une époque où l’on parlait de sang impur… Cette question est extrêmement importante, et je crois que ce qui fonde la République, c’est de concevoir le droit du sol comme une citoyenneté politique. Très

Cela n’a strictement rien à voir avec la République : nous étions dans une période de grande faiblesse démographique par rapport à l’Allemagne et le législateur s’est

Ce texte est destiné à lutter contre les étrangers qui entrent en France de manière irrégulière et qui voudraient y rester bien qu’ils n’y aient pas droit. Là, nous avons affaire à des enfants qui sont en France en situation régulière, qui doivent « faire nation » avec nous, et vous leur fermez la porte. En fait, vous fabriquez des gens extérieurs à la nation française. Nous n’avons vraiment pas la même conception de ce que veut dire « faire nation

Dès que le peuple français a eu la possibilité de s’exprimer, il a inscrit le droit du sol parmi les fondements de notre nation. À la Révolution, tout homme ayant vécu un an sur notre territoire a reçu la possibilité de devenir Français. Pourquoi ? Parce que la France s’est constituée comme une nation politique,

– « que s’agissant d’une telle condition mise à l’acquisition de la nationalité française par l’effet de la naissance sur le territoire français, » – le droit du sol – « il était loisible au législateur

C’est un fait historique ! J’ai le droit d’être d’accord avec lui ! À l’origine, disais je, le droit du sol a été créé pour une raison simple : faire face à la poussée démographique allemande et rendre nos armées capables de mettre autant d’hommes que possible sur le front en cas de mobilisation générale.

mais une vague idée. Je rappelle qu’en 2016, selon l’Ifop, 47 % des lycéens français musulmans plaçaient la charia au dessus des lois de la République.

abject ! Cela, les Français l’ont parfaitement compris, mes chers collègues. C’est à vous de l’admettre enfin : la suppression de cette stupide loi du sol est autant une évidence qu’une urgence

de l’immigration : 210 940 personnes en 2014, 250 000 en 2015, 242 000 en 2017, 250 550 en 2018, 276 600 en 2019, 315 000 en 2022,

Les conditions d’accès à la nationalité, notamment pour les mineurs, restent relativement favorables, ce qui est susceptible de renforcer l’attractivité du territoire français. Aussi, en commission des lois, nous avons souhaité resserrer ces conditions pour les mineurs étrangers nés en France de parents étrangers.

rectifié de M. Ravier ne peut qu’être écarté, puisqu’il est manifestement inconstitutionnel.

et intolérable. Comparer, dans un débat sur le droit du sol, des êtres humains à des animaux n’est pas acceptable, quelle que soit

Ce n’est pas d’une grande élégance, je le reconnais, mais nous sommes tous ravalés au rang de bêtes dans cette histoire. Ce qui me heurte le plus dans ce propos, c’est que la métaphore employée

a privé de liberté syndicale, professionnelle, religieuse, de toutes les libertés fondamentales, des millions d’individus ! Monsieur Gay, vous devriez vous faire plus modeste, plus discret…

Le scrutin est ouvert.

L’assimilation resterait ainsi présumée, à la différence du régime de la naturalisation, mais l’État aurait la possibilité d’apporter la preuve de la non assimilation et de s’opposer à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Quel est l’avis de la commission

commission. Cet amendement tend à prévoir une condition d’assimilation préalable à l’acquisition de la nationalité par le droit du sol. Une telle condition existe déjà pour l’acquisition de la nationalité par naturalisation.

tendant à adapter aux caractéristiques et contraintes particulières de Mayotte les règles d’acquisition de la nationalité française par une personne née en France de parents étrangers, le Conseil d’État avait recommandé que soit menée une campagne d’information, à Mayotte et à destination des pays d’origine des personnes y immigrant irrégulièrement, sur l’état du droit qui résulterait du vote de ce texte. Les dispositions de cette proposition de loi ont finalement été intégrées dans la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

pour faire connaître l’état du droit aux femmes et aux hommes, français ou étrangers, en situation régulière, qui seraient tentés de reconnaître des enfants qui ne sont pas les leurs. Nombreux sont ceux qui ignorent les peines

Par ailleurs, cette infraction a des conséquences patrimoniales importantes, puisqu’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants reconnus pourrait être demandée par la mère et des droits sur l’héritage pourraient être accordés à des enfants. Il est bien sûr indispensable d’accentuer en aval la lutte contre ces comportements délictueux.

au droit du sol. Un article du code civil empêche déjà l’acquisition de la nationalité par toute personne condamnée à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis. Néanmoins, cet article ne s’applique pas aux enfants nés de parents étrangers

empêcher un enfant né sur le territoire français, y ayant vécu jusqu’à l’âge de 18 ans, parce qu’il a été condamné à une peine de six mois d’emprisonnement, d’acquérir la nationalité française jusqu’à la fin de sa vie.

La réflexion sur la question de la nationalité est essentielle pour notre pays. La nationalité est un pilier fondamental de l’identité de notre nation. Il est impératif que notre législation reflète les valeurs et les intérêts de la France. Être Français s’hérite ou se mérite. Ainsi l’amendement que nous vous soumettons aujourd’hui est une première étape vers l’alignement de notre législation sur cette vision. Le droit du sol tel qu’il est actuellement consacré accorde automatiquement la nationalité française, à sa majorité, à toute personne née sur le territoire français, quels que soient ses antécédents familiaux. De même, le double droit du sol permet à un enfant, né en France de parents étrangers, d’acquérir automatiquement la nationalité française. Bien que ces principes aient leur légitimité, ils doivent être revus pour s’assurer qu’ils correspondent aux intérêts et aux valeurs de notre nation. La réforme constitutionnelle proposée durant la campagne présidentielle par Marine Le Pen a pour objectif de redéfinir les critères de la nationalité française, notamment en fixant des conditions plus strictes pour son acquisition. Dans cette optique, il est logique de commencer dès à présent à supprimer les dispositions législatives qui s’opposent à cette vision en éliminant les articles de notre législation consacrant le droit du sol et le double droit du sol. Nous enverrions ainsi le signal fort que la nationalité française ne peut être octroyée automatiquement, mais qu’elle doit être gagnée par des actes et des engagements envers notre nation.

au cours ou à l’occasion d’un engagement opérationnel et qui en fait la demande », ou, en cas de décès de l’intéressé, à ses enfants. Cette disposition illustrait une réalité de nombreux étrangers œuvrent quotidiennement au service de la France, sous les drapeaux, mais aussi dans la vie civile. Le Gouvernement a ainsi à sa main diverses dispositions juridiques permettant d’octroyer la nationalité française à des personnalités étrangères

l’amendement n° 346 rectifié . Cet amendement tend à allonger le délai de résidence au terme duquel la naturalisation peut être accordée à l’étranger résidant habituellement en France,

De plus, les personnes étrangères font l’objet d’un accueil incomparablement plus généreux en France que partout ailleurs, qu’il s’agisse des réfugiés, des demandeurs d’asile, des mineurs isolés ou encore des étrangers en situation irrégulière. La parole

une communauté de destin. À cela, on ne saurait prétendre à la légère. C’est pourquoi le critère de résidence de cinq ans ne semble pas suffisant. De même qu’un pays peut assimiler des individus, mais pas des masses, il peut assimiler sur le temps long, mais pas dans la précipitation.

là ne ferait qu’aggraver la crise civique et les fractures de la société. Ce serait nier ce qu’est la France, nier ce que veut dire être Français. de mettre un terme à la déconstruction juridique des mots et du sens des choses, car il y a bien une culture et une identité françaises. Ceux qui disent le contraire participent au wokisme qui ronge notre État et notre civilisation.

D’un côté, il est important de reconnaître que de nombreuses personnes peuvent entretenir des liens culturels, familiaux ou professionnels avec plus d’un pays. De l’autre, la binationalité ou la multinationalité peut susciter des questions en matière de loyauté et de cohésion nationale, comme en attestent les événements récents qu’a traversés notre pays.

ainsi qu’à renforcer le lien entre la nationalité et la loyauté envers la France. Nous défendons en effet depuis toujours le principe de l’assimilation. Acquérir la nationalité française, c’est épouser les valeurs et l’histoire françaises ; devenir Français est un acte d’amour. Comme tel, il semble légitime qu’il soit unique. Faire Nation est un plébiscite de chaque jour. Si le désir d’un étranger est de devenir Français, il serait anormal qu’il conserve la nationalité du pays qu’il a volontairement quitté. Cependant, notre proposition est placée sous le signe du pragmatisme. À ce titre, elle intègre la possibilité d’accords bilatéraux négociés au cas par cas

de nombreuses personnes sont traversées de liens transnationaux. Pour toutes ces raisons, nous défendons avec vigueur le principe de la suppression de la binationalité, tout en laissant à nos services diplomatiques – fort malmenés depuis six ans – le soin de construire des accords au cas par cas selon les intérêts de la France. Quel

Cet amendement vise donc à déchoir tous les binationaux, fussent ils nés Français, de leur nationalité s’ils affichent clairement une allégeance habituelle et manifeste à une autre nation contre la France, son peuple et ses règles.

a validé en 2020 le principe de la déchéance de nationalité pour les terroristes. Il est urgent de l’étendre à ceux qui terrorisent les Français au quotidien, qui leur rendent la vie impossible en tuant, en pillant, en frappant, en dealant, en violant, en volant nos compatriotes. Je m’en remets à l’analyse de Robert Badinter, apprécié sur ces travées, qui a, lui aussi, défendu la déchéance de nationalité

connu et reconnu. La Nation est une famille, nous ne sommes pas tenus de garder à nos côtés les pièces rapportées qui déchirent notre contrat social et moral, notre pacte civil, notre fraternité, notre identité, notre réputation. vous qui a inventé le principe de la déchéance de nationalité ? Un certain Raymond Poincaré, en 1927. Savez vous qui était son ministre de l’intérieur ? Un certain Albert Sarraut, radical socialiste. Savez vous qui a mis en place le principe de la déchéance de nationalité pour les naturalisés Français

III République. Certes, elle avait bien des défauts, mais elle n’a jamais failli sur un point : la Nation. Vous connaissez les mots d’Ernest Renan : « Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une, constituent cette âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre dans le présent. L’une est la possession en commun d’un riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage qu’on a reçu L’intégration, c’est le simple fait de vivre ensemble ; l’assimilation, c’est devenir une partie de la Nation. L’intégration, c’est la vie en colocation ; l’assimilation, c’est l’appartenance à une même famille. Dans une colocation, la vie commune est passagère, transitoire et déterminée dans le temps

L’assimilation n’est pas l’oubli de soi, c’est la rencontre et la fusion avec l’autre, ce corps qui vous accueille quand bien même vous lui fûtes étranger, qui vous aime et qui vous soutient, pour peu que vous remplissiez vos devoirs à son égard. Être Français n’est pas seulement un droit, c’est une somme de devoirs à accomplir pour en être digne. En remplaçant « intégration » par « assimilation », vous participerez, mes chers collègues, à faire briller davantage ce si beau mot : Français.

notion centrale de notre programme plébiscité par 13 millions de Français à la dernière élection présidentielle. La priorité nationale est la contrepartie logique et naturelle à la nationalité. En effet, les Français doivent bénéficier d’un droit prioritaire – et non exclusif – chez eux dans l’accès au logement social, aux aides sociales ou à l’emploi. Ainsi, il ne s’agit en rien d’une disposition de discrimination ou d’exclusion, mais c’est bien un droit logique et nécessaire, appliqué dans 95 % des

Pourtant, ce brave ministre radical socialiste a soutenu au mois de décembre 1931 une loi instaurant la préférence nationale à l’emploi en période de forte crise économique. Heureusement que je suis là pour remettre à l’honneur le radical socialisme La priorité nationale ou la préférence nationale – appelez cela comme vous le souhaitez – n’est pas une exception. Elle est la règle dans la plupart des pays du monde, au premier rang desquels les États Unis ou le Brésil de Lula.

Notre pays compte 5 millions de chômeurs. Tout doit être mis en œuvre pour les aider à retrouver un emploi. J’ai bien conscience que la priorité nationale n’est pas une recette miracle, mais elle aidera quelques centaines de milliers de Français à retourner au travail. Quand bien même un seul d’entre eux serait concerné, ce résultat me réjouirait. Retrouver un emploi, c’est retrouver la dignité, la fierté, le chemin de la vie sociale. La Nation consiste à prendre d’abord soin des nôtres, des Français, trop souvent soumis à une concurrence étrangère déloyale, qui coûte moins cher, qui réclame moins, qui ne s’organise pas.

plutôt que d’employer des Français qui connaissent le droit du travail. Je préfère protéger le salarié français que l’immigré sans papiers et cette position ne souffre d’aucune ambiguïté ni d’aucune hésitation. Il y a trente ans déjà, je préférais mes filles à mes cousines, mes cousines à mes voisines et mes voisines aux étrangères. Maintenant que j’ai deux filles, vous comprendrez que je tienne à cette priorité ! Mes chers collègues, je vous invite donc à voter cet amendement de bon sens.

ont décidé de laisser sans réponse les demandes de rendez vous pour régularisation de travailleurs, enterrant de fait la circulaire sur leur territoire. Face à la pénurie de moyens humains, les renouvellements de titres de séjour sont en effet privilégiés dans de nombreuses préfectures. L’article 3 du projet de loi, y en aura une à l’issue de nos travaux, prévoit dans tous les cas la mise en place expérimentale d’un nouveau titre de séjour de plein droit. Nous estimons que cette expérimentation ne peut être évaluée correctement sans la remise au Parlement d’un rapport sur la mise en œuvre et les limites de la circulaire Valls au regard des enjeux socioéconomiques de nos territoires. Quel est l’avis de la

pour un rappel au règlement.

Ils demandent ce que la raison et la justice voudraient que nous demandions, à savoir la régularisation de tous les travailleurs sans papiers. L’article 3, qui reçoit tant de critiques sur les travées de la droite, réduit pourtant toujours ces travailleurs, dont une grande partie exercent des métiers difficiles et dangereux, à l’immigration

Comme le constate Émeline Zougbédé, sociologue au CNRS, la liste des métiers en tension telle qu’elle existe aujourd’hui ne correspond pas du tout aux postes qu’occupent les sans papiers. Problème, que faites vous des travailleurs sans papiers qui ne sont pas employés dans les prétendus métiers en tension ? Que ferez vous de ceux qui le sont, puis qui ne le seront plus et de ceux qui travaillent depuis des années et font tenir des entreprises et des secteurs entiers, participant ainsi à l’effort collectif ? la position raisonnable et humaniste, c’est la régularisation de tous les travailleurs sans papiers, de plein droit, par l’octroi d’un titre de séjour durable. Nous en sommes loin ! Même limitée aux emplois vacants, la droite trouve qu’une telle disposition est encore trop, par pure idéologie

la carte de séjour temporaire mention “travail dans des métiers en tension” relèverait de la seule initiative du travailleur étranger. Elle serait délivrée de plein droit sous réserve de la preuve, apportée par tout moyen, d’une ancienneté de résidence sur le territoire

chers collègues, régulariser une personne qui vit en France, qui y travaille, c’est tout simplement reconnaître sa participation à la vie de notre société.

Encore une fois, nous ne comprenons pas du tout l’effervescence suscitée par cette disposition sur les métiers en tension. Fallait il créer un nouveau titre de séjour avec des critères ouvrant un droit à régularisation dans les métiers en tension ? Non. n’est pas nouvelle, c’est ce que nous répétons depuis des mois. Notre ligne sur le sujet est parfaitement claire et n’a pas bougé : le plus efficace

Nous sommes attachés au fond de cet article, pas à sa forme. Comme nous le souhaitons, le dispositif proposé prévoit bien de modifier le régime applicable en matière d’autorisation de travail. Comme cela a été rappelé, un salarié sans papiers qui souhaite régulariser sa situation

moi d’exprimer les regrets du groupe CRCE K. Nous n’avons jamais considéré que l’article 3 était une panacée. Nous avions plein de propositions à formuler pour en améliorer la rédaction et en étendre l’application.

pas un expert, pas un chef d’entreprise, pas un syndicaliste ne confirme. L’immigration serait incontrôlable. C’est faux ! Aucune statistique ne le valide. Il faudrait revenir sur la dignité des personnes, attaquer les étudiants, refuser de soigner les immigrés. Il faudrait limiter les mariages mixtes et le regroupement familial. C’est ainsi que l’on répondrait à un enjeu de société.

n’ignore ici que notre société ne fonctionnerait pas sans ces dizaines de milliers de travailleurs sans papiers.

Pardonnez moi, mes chers collègues, mais je trouve les postures accusatoires et moralisatrices parfaitement déplacées. Que ceux qui défendent l’idée que la fraude peut être créatrice de droits ne revendiquent pas pour leur compte la morale et ne nous accusent pas d’hypocrisie. Par ailleurs,

C’est la solution de la résignation à ne rien faire pour que les emplois disponibles soient pourvus soit par des Français, soit par des étrangers en situation régulière. Enfin, nous ne pouvons absolument pas

telle mesure nous paraît totalement insoutenable. Que des régularisations soient possibles par l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’État, pour récompenser des conduites exceptionnellement vertueuses et pour permettre

sur l’article. L’article 3 est mort, vive l’article 3 ! Voilà donc le résultat des tractations de la journée. Si l’amendement que la majorité sénatoriale présentera tout à l’heure vise à limiter à la marge la scandaleuse campagne de régularisation massive que proposait le Gouvernement, il ne réglera en rien le problème principal, qui est

2 millions de chômeurs et 3 millions de sous employés, l’économie française peut répondre sans immigration à cette prétendue crise de main d’œuvre qui n’est qu’une crise des salaires et des conditions de travail. Ne vous en déplaise, les Français ne sont pas des fainéants, mais ils ne peuvent continuer à exercer des métiers difficiles pour des salaires de misère à des dizaines de kilomètres de chez eux, alors que le coût de l’énergie et des carburants

des pratiques condamnables au premier sens du terme, puisqu’elles sont illégales. La gauche continue de constituer son armée de réserve électorale, la même que Marx appelait l’armée de réserve du capitalisme, puisque c’est le dumping social qui s’organise avec une pression à la baisse sur les salaires.

d’un article paru hier dans : « Au moment où l’examen du projet de loi sur l’immigration, qui prévoit la régularisation sous conditions des étrangers irréguliers dans les métiers en tension, a démarré en plénière au Sénat, l’étude apporte sa contribution au débat : elle juge que la France gagnerait à s’ouvrir davantage aux minorités et aux immigrants. Des pays comme le Canada ou Singapour ont su gérer le sujet de l’immigration

voiture gouvernementale. Avec l’article 3, elle marquait un virage à gauche, après tous les virages à droite que nous avons connus ; or vous semblez vouloir tourner aussi à droite dans ce virage qui part à gauche. Faites attention, car vous risqueriez de conduire le Gouvernement et la France à droite, non pas vers M. Ravier, mais dans les graviers. Ce serait un déshonneur pour la France.

sur le caractère automatique du titre de séjour accordé dans le cadre de l’article 3 : il aurait alors suffi de justifier que l’on voulait un travail ou d’expliquer que l’on avait un travail, sans vérification de la réalité de celui ci auprès de l’employeur,

mais sur la base de la vérité ! L’ordre du jour appelle la désignation des trente sept membres du groupe de travail préfigurant la commission spéciale chargée d’examiner, sous réserve de son dépôt, le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière et en matière agricole. En application de l’article 8, alinéas 2 et 3, de notre règlement, les listes des candidats présentés par les groupes ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence ne reçoit pas d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement. Il appartiendra au Sénat de transformer ce groupe de travail en commission spéciale, après le dépôt du projet de loi, conformément à l’article 16 de